madame la présidente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

revient sur la question des pénuries de médicaments. Le renforcement de notre souveraineté sanitaire et la relocalisation en France ou en Europe de certains produits de santé ne constituent qu'une réponse partielle à la problématique des pénuries

prendre en compte les surcoûts occasionnés. Cette possibilité de revalorisation de prix doit concerner essentiellement les médicaments pour lesquels une interruption de traitement représente une perte de chance importante pour les patients, ce qui est souvent le cas.

soulignait que la baisse du prix des médicaments originaux, conjuguée à l'augmentation des coûts de production, entraînait un « effet ciseau » pour les industriels, qui préféraient se désengager ou délocaliser hors d'Europe la production des médicaments.

comme ce fut le cas en France jusqu'en 1959. Concernant les brevets qui tombent dans le domaine public, il nous semble indispensable de doter une pharmacie nationale des médicaments et des produits de santé. Le renforcement de notre souveraineté sanitaire et la relocalisation en France ou en Europe de la production de certains produits de santé ne constituent qu'une réponse partielle à la problématique des pénuries qui préexistait à la crise du covid-19. L'amendement n° 505 rectifié,

confirme la tendance observée ces dernières années, qui consiste à baisser le prix des médicaments remboursables originaux ayant perdu leur brevet. En 2018, le rapport de la mission d'information sénatoriale sur la pénurie de médicaments et de vaccins soulignait la baisse du prix

Cet amendement vise donc à prendre en compte l'implantation des sites de production et leur ancienneté, ainsi que le maintien ou l'orientation de nouveaux investissements de l'entreprise sur le sol national, à la fois dans la fixation et la révision des prix par le comité économique des produits de santé (CEPS), afin de limiter les risques de pénuries, de garantir l'accès aux traitements du quotidien et de favoriser la relocalisation de la production des principes actifs les plus critiques.

uniquement en compte dans la fixation du prix des produits de santé l'implantation des sites de production et leur ancienneté, ainsi que le maintien ou l'orientation de nouveaux investissements de l'entreprise. L'amendement n° 690

trop faibles. Entre 2008 et 2019, le nombre de médicaments concernés par une rupture ou un risque de rupture signalés à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé En 2020, l'ANSM évalue le nombre de médicaments en rupture à 2 446. Un quart des Français auraient déjà été confrontés à un refus de délivrance de leur traitement pour cause de pénurie. Selon une étude de la Ligue contre le cancer, 74 % des professionnels ont été confrontés à des pénuries de médicaments contre le cancer. Le renforcement de notre souveraineté sanitaire et la relocalisation en France ou en Europe de la production de certains produits de santé doivent ainsi être de la sécurité sociale pour 2022 sont insuffisantes. Les politiques de relocalisation de la production doivent prendre en compte les coûts découlant de ce type de production. selon l'ANSM, les pénuries concernent principalement des produits anciens, dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Cette prise en compte concerne essentiellement les médicaments pour lesquels une interruption de traitement représente une perte de chance

Aussi, alors que ce dispositif pourrait faire naître des contentieux, cet amendement vise à renforcer son encadrement réglementaire et, partant, sa sécurité juridique. Il prévoit ainsi la définition de critères par décret en Conseil d'État, ce décret étant également chargé de définir les modalités d'engagement et de suivi. J'ai entendu certains collègues ou industriels considérer que l'adoption de cet amendement serait une source de retard pour l'entrée en application du dispositif, voire, ai-je pu lire, un signe de défiance à l'égard du CEPS. Je tiens à rassurer tout le monde : nous n'exprimons aucune défiance envers le CEPS et la commission n'a formulé cette proposition

établir sa doctrine au fil de ses rapports d'activité, ce qui prendra du temps. L'intention de la commission est donc bien d'éviter des contentieux, de sécuriser le dispositif et les décisions du CPES, par un gain en transparence pour le CPES, mais aussi pour l'ensemble des industriels. En effet, croyez bien que les

entre le CEPS et le LEEM. Or cet accord ne limite pas la prise en compte des investissements aux seules capacités de production, mais intègre également les activités liées à la recherche et développement (R&D), et au développement de solutions numériques. En réintégrant ces activités, cet amendement vise donc à rétablir la cohérence de l'article 38 avec les principes qui ont guidé à la signature de l'accord-cadre, réaffirmés par le Président de la République lors du dernier conseil stratégique des industries de santé

En réalité, comme Sanofi, pour optimiser leurs profits, les entreprises sous-traitent l'essentiel de leur recherche médicale auprès d'un réseau de start-up, véritables têtes chercheuses, avec, éventuellement, un rachat Si ce système permet d'optimiser les coûts, grâce aussi au crédit d'impôt recherche (CIR), et de maximiser les bénéfices, le prix, lui, n'en tient guère compte. Cela n'empêche pas Sanofi d'obtenir par exemple un nouveau plan d'investissements publics du Gouvernement, à hauteur de 7 milliards d'euros. Le contribuable et l'assuré payent ainsi deux fois.

dans l'établissement du prix de vente au public de chacun des médicaments fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation parallèle du médicament ou l'entreprise assurant la distribution parallèle du médicament et le comité économique des produits de santé. Ce critère supplémentaire favorisera l'accès précoce des patients aux traitements innovants, l'implantation de centres de recherche ainsi que

Si cette dimension est essentielle pour renforcer l'indépendance sanitaire de l'Europe et de la France, il ne faut pas négliger pour autant les investissements en matière de recherche clinique qui, s'ils sont réalisés en Europe, ont des effets vertueux sur l'ensemble des pays européens, notamment la France. En effet, la recherche clinique permet aux patients d'accéder plus rapidement à des traitements innovants et d'améliorer la pratique des médecins. Plus généralement, elle contribue au rayonnement du système dans son ensemble.

Favoriser le développement des essais cliniques en Europe, c'est donc contribuer à construire un modèle vertueux tant pour les patients que pour le système dans son ensemble et pour le développement économique. La France doit jouer un rôle moteur sur ce sujet l'ambition de faire de notre pays le leader en Europe des essais cliniques figure parmi les annonces phares du Président de la République au conseil stratégique des industries de santé. Afin d'accélérer le développement de la recherche clinique sur le continent européen, cet amendement vise à inclure dans les critères de fixation des prix des produits de santé les investissements

Toute une série de critères ont été évoqués, avec, parfois, une part de pertinence que je ne nie pas, mais, parfois aussi, des lacunes. Oui, il faut soutenir les investissements. Oui, il faut mieux prendre en compte la recherche. Oui, il faut valoriser l'implantation en Europe. Oui, l'empreinte sociale et l'empreinte environnementale méritent aussi d'être prises en considération. Je m'interroge sur les limitations réclamées par les auteurs de certains amendements aux seuls médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Cela ne semble pas opportun. Je m'interroge aussi sur la prise en compte particulière des solutions numériques facilement délocalisables. Par ailleurs, certains évoquent les seuls coûts supplémentaires. Pourquoi pas, mais comment les estimer ? Si l'intention est louable, en réalité, la portée opérationnelle n'est pas tenable et c'est donc tuer dans l'oeuf cet objectif de soutien industriel.

Je rappelle que cet article n'est pas le seul outil au service d'un soutien à l'industrie des produits de santé. L'accord-cadre du CEPS et du LEEM offre une palette de mesures avec des engagements de stabilité des prix, notamment au regard des investissements qu'il faut valoriser. Il me semble- c'est la position de la commission depuis le début -qu'il faut conserver une rédaction simple et efficace pour cet article et qu'il appartiendra au CEPS et au Gouvernement de préciser le ciblage, les modalités et critères de prise en compte des facteurs industriels.

le contexte. La crise du covid-19 a mis en lumière l'insuffisance des capacités de production nationales et européennes face aux pics de demandes pour certains médicaments et dispositifs médicaux essentiels. Accentuée par la fermeture des des frontières nationales, elle a ainsi révélé la dépendance de l'industrie française et européenne, en matière tant de principes actifs que de dispositifs médicaux fabriqués hors d'Europe. Par conséquent, dans un objectif de sécurité d'approvisionnement et pour inciter

dans la fixation des prix des produits de santé. Dans l'objectif d'accroître les capacités de production et, ainsi, de limiter les risques de rupture d'approvisionnement, cette mesure propose d'inscrire un nouveau critère de fixation des prix de produits de santé, donc de tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation

ainsi que l'implantation des sites de production de production dans les critères de fixation de prix. Là aussi, pourquoi limiter la prise en compte de la relocalisation dans la fixation du prix ? Il peut y avoir aussi des besoins sur des produits qui ne sont pas anciens.

Cela ne nous semble pas avoir une incidence sur la relocalisation des industries, en tout cas sur la fixation du prix qui doit en résulter. Qui plus est, dans le cadre d'accords qui existent déjà, ce sont

prévoit déjà la valorisation des investissements réalisés ou à venir, et précise les conditions dans lesquelles certains produits peuvent être éligibles à la hausse des prix en cas de risques importants pouvant impacter la production et la commercialisation. La valorisation des investissements réalisés ou à venir est donc déjà prise en

des sites de production. C'est une garantie que de les avoir sur place. Je souhaite toutefois ajouter un critère, qui prend en compte la politique industrielle,

de marquer notre indépendance sanitaire dans le domaine de production de principes actifs, de médicaments ou de dispositifs médicaux. Nous sommes passés en dix ans de la première à la quatrième place parmi les producteurs européens de médicaments, ce qui n'est pas satisfaisant. Nous faisons face à une importante politique de régulation des prix et la politique de régulation comptable menace de réduire encore notre souveraineté sanitaire, sanitaire, tant par la délocalisation des usines de production que par l'absence d'installation de ces dernières en France. Quand on parle des usines de production, on parle également de la sous-traitance ou des façonniers Au-delà du plan gouvernemental, qui prévoit notamment la relocalisation de la production de principes actifs- comme le paracétamol -sur le territoire national, avec l'objectif de produire, conditionner et distribuer ce médicament d'ici à trois ans

mets aux voix l'amendement n° 272 rectifié. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

si l'enjeu est de valoriser à la fois la relocalisation et l'innovation, ces entreprises remplissent tous les critères. Elles jouent un rôle primordial dans l'accès des patients français aux médicaments innovants, souvent dans des cas où il n'existe pas d'alternative efficace. Mais pour ces laboratoires, l'implantation de sites de production n'arrive que dans un second temps, après qu'ils se sont assurés, pour leur viabilité, que le prix fixé pour le premier traitement commercialisé permet à la filiale de développer son activité en France. Nous proposons donc que la situation particulière des biotech soit prise en compte dans la fixation du prix du médicament avec le CEPS.

à Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à renforcer la transparence de l'ensemble des informations transmises par l'entreprise pharmaceutique au comité économique des produits de santé, en intégrant dans la liste les critères de fixation des prix des médicaments,

Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France. En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis 2017, il n'existe pas d'obligation de révision des prix. Par cet amendement, nous défendons l'idée que le prix de vente d'un médicament doit être révisé à un niveau inférieur ou abaissé par convention ou, à défaut, par une décision du CEPS dans trois cas : après cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie des prix au niveau

est l'avis de la commission ? Des mécanismes de révision à la baisse sont déjà prévus dans le code de la sécurité sociale. Ces baisses se font par convention entre le CEPS et les industriels à défaut d'accord, le CEPS les décide de manière unilatérale. Ces fixations de prix à un niveau inférieur ou révisions à la baisse s'appuient sur une série de critères, notamment d'ancienneté ou de comparaison de prix, selon les canaux d'achat ou selon les prix pratiqués à l'étranger, par exemple.

de lutter contre une dynamique d'inflation des prix des médicaments qui ne serait pas justifiée. Valeur thérapeutique et apport clinique pour le patient doivent rester évidemment les principaux critères de tarification des médicaments. Il peut arriver que la Haute Autorité de santé réévalue cet apport clinique au regard de données en vie réelle. de données en vie réelle. Une amélioration du service médical rendu, dans le système que vous proposez, si l'on adoptait cet amendement, ne pourrait plus être prise en compte.

sur le marché d'un médicament. Il vise à répondre aux interrogations relatives à la transparence du prix des médicaments qui s'expriment en matière de démocratie sanitaire et sont régulièrement relayées par nos concitoyens.

une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficile la distinction entre la part des investissements publics et celle des investissements privés. Il est donc souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d'un médicament. Cet amendement oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements de recherche et développement dont ils ont bénéficié lors du développement d'un médicament. Le CEPS, qui sera destinataire de cette information, pourra en tenir compte lors de ses négociations sur la fixation des prix avec les industriels. Toutefois, nous avons bien conscience que retracer précisément les effets des différentes sources d'investissement public sur le développement d'un médicament soulève de nombreuses questions pratiques. C'est la raison pour laquelle un décret d'application viendra préciser les conditions de mise en oeuvre de cet article au plus tard le 1 janvier 2023.

distinguable la part respective des investissements publics et privés dans le développement d'une nouvelle molécule. La transparence est un enjeu important d'un point de vue non seulement économique, mais également démocratique. Notre amendement vise à isoler le montant des investissements publics de recherche bénéficiant aux entreprises pour l'élaboration de nouveaux médicaments tant sur la généalogie des molécules, à travers les déclarations par les industriels d'éventuels rachats de brevets ou d'entreprises leur ayant permis d'obtenir leur droit de commercialisation, que sur la nature des investissements publics incluant exonération d'impôts ou de cotisations.

Enfin, il s'agit d'obtenir les données médicament par médicament, dans un format adapté à des négociations de prix conduites pour chaque produit, car leur lisibilité ne peut pas être dissociée de l'impératif de transparence qui motive notre amendement.

de distributeurs au détail de produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables de déclarer au comité économique des produits de santé le prix de vente, le cas échéant au distributeur au détail, de chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur. Les fabricants de montures optiques se retrouvent soumis à cette obligation de déclaration de tous leurs prix de vente du simple fait que leurs produits sont des dispositifs médicaux, alors même que les prix de vente des montures optiques ne sont pas négociés avec le CEPS.

nous semble pas aller dans la bonne direction. Je vous le rappelle, la mesure de déclaration de prix est la conséquence directe de recommandations de plusieurs rapports récents relatifs à la régulation du secteur des dispositifs médicaux et de prestations associées. Ceux-ci insistent sur la nécessité pour le CEPS de disposer de plus d'informations sur le secteur qu'il est chargé de réguler. Il existe en effet une asymétrie d'information entre le comité et les entreprises avec lesquelles il négocie, ce qui rend l'exercice de négociations très difficile. Ainsi, toutes ces informations sont nécessaires pour objectiver les secteurs pouvant faire l'objet de révisions tarifaires, ainsi que les économies susceptibles d'être réalisées. Elles sont donc utiles,

alors que les besoins progressaient durant les périodes de pic de la pandémie de la covid-19. Les salariés de l'Établissement français du sang étaient en grève le 21 octobre dernier, car ils font partie des « oubliés du Ségur de la santé Après des suppressions massives de postes ces dernières années, et alors que les problèmes de recrutement sont extrêmement importants- je crois que l'on parle de 300 postes vacants -, les personnels de cet établissement assurant une mission publique demandent à pouvoir bénéficier de la revalorisation salariale du Ségur de la santé en raison de leur appartenance au secteur privé non lucratif, en première ligne durant la crise sanitaire. Notre amendement a pour objet- nous ne pouvons pas aller plus loin compte tenu de l'article 40 de la Constitution -la remise d'un rapport sur la manière de restructurer la filière française

ont déjà été soulignées, je crois, par le ministre Olivier Véran. Des travaux sont en cours avec l'ensemble des parties prenantes pour apporter des réponses vraiment structurelles à l'approvisionnement des patients français dans ces produits essentiels et spécifiques. Je vous rappelle les trois axes de travail qui ont été définis dans ce cadre

de la filière française du plasma que sont, d'une part, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et, d'autre part, bien entendu, l'Établissement français du sang. Le Gouvernement rendra publics et mettra en oeuvre les axes opérationnels issus de ces travaux

à Mme Émilienne Poumirol. Cet amendement vise à supprimer l'article 38 , qui a pour objet d'expérimenter la prise en charge du sevrage tabagique par les substituts nicotiniques lorsqu'ils sont dispensés par les pharmaciens d'officines sans ordonnance. telle mesure semble viser une nouvelle fois à pallier le manque de médecins sur notre territoire. À notre sens, il n'est pas raisonnable de démédicaliser le sevrage tabagique. La consultation antitabac n'est pas une simple prescription de ou de gomme. De plus, l'idée selon laquelle le prescripteur serait aussi le vendeur est contraire à un principe fondamental de médecine, avec un risque de dérive. Nous avons pu l'observer pour les examens radiologiques, en nette progression depuis que les radiologues sont autorisés à prescrire eux-mêmes les examens qu'ils peuvent pratiquer.

l'avis de la commission ? En permettant la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques délivrés sans ordonnance en officine, l'expérimentation

Cependant, certains éditeurs de logiciels n'ont toujours pas adapté leur outil à la législation. Les pharmaciens ne peuvent donc pas se soumettre à une telle obligation. Cette éventualité doit être envisagée par le législateur, et des pénalités financières doivent s'appliquer aux éditeurs de logiciels non conformes.

de leur éditeur de logiciel pour adapter le logiciel et leur permettre de se connecter aisément au répertoire national de vérification des médicaments. Toutefois, l'article 39 prévoit bien

et indiquer ainsi qu'il a demandé à l'éditeur d'adapter en conséquence son logiciel d'aide à la dispensation. Je pense que les éditeurs de logiciels n'ayant pas fait évoluer leur système sont connus des autorités. Et la procédure contradictoire permettra aux pharmaciens d'officine qui ne pourraient

Mais la méthode du Gouvernement est critiquable à un double titre. D'abord, les mesures en question ont trait aux conditions d'exercice des professionnels de santé. Or le Conseil constitutionnel a déjà considéré par le passé que de telles dispositions n'avaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale si leur incidence directe sur l'équilibre des comptes sociaux n'était pas établie. Le Gouvernement est donc directement responsable de cette entorse au champ organique des lois de financement de la sécurité sociale, et l'Assemblée nationale n'a pas manqué de s'engouffrer dans la brèche en introduisant plusieurs articles additionnels. additionnels. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous est transmis contient pas moins de six articles organisant un accès direct à différentes professions de santé, la plupart par voie d'expérimentation. Or aucune de ces dispositions n'a fait l'objet d'une concertation avec les représentants des professionnels concernés.

Or supprimer l'étape de la consultation médicale préalable n'est pas nécessairement la clé d'un accès optimal aux soins. Faciliter l'accès aux soins, d'accord, mais pas à n'importe quel prix ! La qualité et la pertinence des soins doivent rester cardinales dans l'organisation des parcours. C'est à cette exigence que tendent à répondre les amendements proposés par la commission

Nos concitoyennes et nos concitoyens ont de plus en plus de difficultés pour obtenir des rendez-vous chez les généralistes ou chez les spécialistes. Nous en sommes toutes et tous conscients ici. Pour rappel, la délégation aux droits des femmes vient de remettre un rapport indiquant que treize départements en France n'ont pas de gynécologue médical. Dès lors, comment gère-t-on la pénurie ? Est-ce une bonne idée de confier certaines missions aux professions paramédicales ? Pour notre part, nous sommes favorables à la reconnaissance des compétences de ces dernières. Mais n'est-ce pas d'abord une façon de gérer la pénurie alors que nous savons pertinemment que le manque de médecins est dû en partie des années de ? Quelles seront les conséquences à long terme ? Ne va-t-on pas assister à une médecine à deux vitesses et créer davantage d'inégalités ? J'en viens plus spécifiquement à l'article 40 Honnêtement, au sein de notre groupe, nous ne savons pas si, d'un point de vue médical, autoriser les orthoptistes à réaliser des bilans visuels, à dépister à dépister chez l'enfant l'amblyopie, à prescrire des lentilles et des verres correcteurs, missions exercées jusqu'ici par des ophtalmologistes, est la bonne solution.

déclare : « Le PLFSS pour 2022 contient des mesures qui morcellent nos exercices et ont été écrites et publiées sans concertation avec les représentants des médecins et des autres professions de santé concernées. [ que nous travaillons actuellement en bonne entente et articulation avec les infirmières, les kinésithérapeutes, les orthoptistes et les sages-femmes. « Loin d'améliorer l'accès aux soins, de tels transferts de tâches non concertés n'agissent pas sur la pénurie des médecins et des soignants. [ ...] Ils fragilisent le périmètre de nos métiers et rendent incompréhensibles les parcours de soins pour les patients, introduisant un doute sur la pertinence des soins. [ ...] « Enfin, ces décisions, prises sur des arguments statistiques et non médicaux, entraînent une dégradation de la qualité des soins, responsable d'une perte de chance pour les patients et de risques juridiques pour les professions nouvellement sollicitées.

Durant le processus d'élaboration du PLFSS, le ministère a indiqué à plusieurs organisations professionnelles de la santé que le texte ne contiendrait aucun élément relatif aux rapports entre les professions de santé dans ce texte.

entre les professions de santé, vous semez la discorde : c'est une erreur.

sur l'article. Mes chers collègues, j'entends les arguments de ceux qui d'entre vous qui souhaitent la suppression de l'article 40. Pour autant, il convient de regarder le bénéfice-risque, dans un contexte de manque d'ophtalmologistes, en particulier dans nombre de départements où les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous sont très longs, souvent de plusieurs mois.

dans deux ou trois ans, si d'éventuelles difficultés devaient être constatées. Je voterai donc contre les amendements visant à supprimer l'article 40.

tout en garantissant une prise en charge sécurisée pour les patients. L'article prévoit un certain nombre de garanties, sur lesquelles je reviendrai. En plus de réduire les délais de rendez-vous, la mesure permettra de recentrer le travail des ophtalmologistes sur le traitement des pathologies oculaires complexes, l'âge (DMLA) ou le glaucome. Pour rappel, les orthoptistes sont des professionnels de santé spécialisés dans le traitement des troubles oculaires. Ils travaillent depuis de nombreuses années en collaboration avec les ophtalmos

En réalité, la mesure dont nous discutons est déjà en vigueur depuis de très nombreuses années, chez l'immense majorité de nos voisins européens. Cette nouvelle compétence d'accès direct favorisera l'installation d'orthoptistes partout en France. Elle contribuera à la lutte contre cette désertification médicale généralisée que nous regrettons, notamment- nous l'espérons -dans les zones sous-denses, où les besoins sont les plus criants. le décret d'application de la mesure sera concerté, là encore, avec l'ensemble des acteurs de la filière. Il tiendra bien évidemment compte des compétences des orthoptistes. Je le répète : nous sommes vraiment convaincus

prescription de lentilles de contact et de lunettes, réalisation d'un bilan visuel, dépistage chez l'enfant de l'amblyopie et troubles de la réfraction. Or les orthoptistes, durant leurs trois années d'études contre douze pour les ophtalmologistes, ne semblent pas s'être correctement préparés à ces nouveaux actes médicaux. Par ailleurs, il semble que les professionnels concernés par ce dispositif, et particulièrement les ophtalmos- médecins prescripteurs, faut-il le rappeler ? -, n'y aient pas été associés ou seulement partiellement. Cela risque à mon sens de

Je présente cet amendement au nom de Mme Joseph. L'amélioration de l'accès aux soins est un objectif salutaire et nécessaire, mais il ne doit pas se faire au détriment des patients. À cet égard, le recours aux orthoptistes pour réaliser une primo-prescription pose plus de difficultés qu'il ne résout de problèmes. Je respecte les orthoptistes, mais ils ne suivent pas la même formation que les ophtalmologues. Ils ne peuvent détecter et gérer les pathologies ophtalmologiques. Une ouverture de la primo-prescription découragerait les ophtalmologues, qui effectuent non seulement de longues études, mais poursuivent également un apprentissage tout aussi long par la suite. Les causes de l'allongement des délais de rendez-vous auprès des ophtalmologues sont à rechercher ailleurs. En outre, les délais se sont récemment raccourcis. D'autres mesures sont à prendre, comme l'encouragement à la création de cabinets dans les zones peu dotées. Enfin, la médecine n'est pas une solution. Nous n'avons pas envie de centres de santé sans scrupules proposant

principalement centrée sur la rééducation visuelle et la réalisation du bilan orthoptique. Ils ne sont formés ni pour l'analyse ni pour le diagnostic de pathologies. Un rendez-vous avec un ophtalmologue, ce n'est pas simplement une commande de paires de lunettes. L'élargissement des prérogatives des orthoptistes pourrait conduire à une dégradation des soins en ophtalmologie. Il faut un médecin pour dépister les maladies, grâce à un examen clinique global. Les ophtalmologues craignent, avec raison d'ailleurs, une résurgence de maladies repérées trop tardivement, avec des risques de cécité et de perte d'autonomie.

pour obtenir un rendez-vous était de 26 jours en 2021, contre 42 jours en 2019, soit une baisse de 38 % sur deux ans,

constitutionnel d'égalité d'accès aux soins. Sur le fondement de cet argument, le Gouvernement propose que les orthoptistes puissent désormais réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs ou des lentilles de contact à un patient, sans que ce dernier ait

d'éventuelles pathologies oculaires « silencieuses », asymptomatiques, à partir d'actes que ne peut réaliser l'orthoptiste. Cela est d'autant plus valable pour la prescription de lentilles de contact. Renoncer aux spécialistes en premier recours, c'est renoncer à la prévention et risquer une dégradation du pronostic, s'il s'avère tardif.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

première consultation auprès d'un ophtalmologiste pour l'entrée dans la filière de santé visuelle. La primo-consultation et la primo-prescription ne peuvent être réalisées, de notre point

sous la prétendue supervision d'un ophtalmologiste référent, des paramédicaux multiplieront les prescriptions de lunettes, au risque d'ailleurs d'un appauvrissement de leur pratique.

entre professionnels pour construire une véritable filière visuelle. Nous craignons qu'elle ne réduise la possibilité pour nos concitoyens d'accéder aux ophtalmologistes pour le diagnostic de certaines maladies. Cet amendement vise donc à encadrer l'intervention des orthoptistes des orthoptistes et à leur octroyer la possibilité, dans une zone dite sous-dotée, déterminée par les ARS, de renouveler une première prescription première prescription médicale sur avis du médecin. Cette solution, j'en conviens, n'est pas idéale, puisqu'elle ne répond pas au manque d'ophtalmologistes dans de nombreux territoires, mais elle permet de répondre à l'urgence que représentent les déserts médicaux, sans mettre en péril la santé de nos concitoyens.

Mme Raymonde Poncet Monge. La prescription de lentilles de contact suppose un examen plus complexe qu'une simple prescription de lunettes. Le législateur lui-même ne s'y est pas trompé puisqu'il s'est écoulé presque dix ans entre le premier décret, en 2007, autorisant les opticiens-lunetiers à renouveler ou adapter les lunettes correctrices après un examen de réfraction, et le second, en 2016, qui a élargi leur périmètre de compétence aux lentilles de contact, pour la limiter aussitôt, puisqu'ils ne peuvent que les renouveler ou les adapter, et non les prescrire. La prescription de lentilles ne peut pas faire l'économie d'un examen approfondi des yeux et d'un dépistage des contre-indications, qui peuvent conduire le spécialiste à les déconseiller pour préconiser l'équipement en lunettes. Nous demandons donc que soit supprimée la disposition de l'article permettant aux orthoptistes la primo-prescription de lentilles de contact.

prévue pour les orthoptistes en la conditionnant au suivi régulier des patients par un médecin ophtalmologue. La fréquence du suivi est adaptée selon l'âge du patient et correspond à la durée de validité d'une prescription de verres correcteurs

de présenter une pathologie qui ne serait pas détectée lors de ces actes. Nous l'avons déjà dit, l'idée est bien de mieux encadrer médicalement cette nouvelle compétence accordée aux orthoptistes. En conséquence, l'amendement prévoit que les textes d'application soient pris après avis du Conseil national professionnel d'ophtalmologie, ce qui nous paraît essentiel. Il est également précisé que les bilans visuels ne concerneront que des patients compris dans une tranche d'âge afin de prévenir les pertes de chance, notamment pour les patients les plus âgés.

qui ont pour objet la surveillance de la croissance et du développement de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que le dépistage des anomalies ou déficiences sensorielles, notamment visuelles et auditives, des troubles du langage et des troubles du comportement. L'article R. 2132-1 du code de la santé publique liste ces examens obligatoires et en organise le calendrier. Il y aura donc redondance d'actes pour le visuel, car le suivi pédiatrique s'intéresse à l'enfant dans sa globalité et tend à éviter le morcellement de la prise en charge. Le risque est l'abandon par les familles de ces examens complets auprès des médecins spécifiquement formés à cet effet. D'autre D'autre part, l'article 40 ne dit rien de la responsabilité de l'orthoptiste dans le cas où il n'aurait pas détecté une pathologie nécessitant une prise en charge médicale rapide. Il paraît dangereux pour la qualité des soins et le dépistage des pathologies oculaires d'autoriser les orthoptistes à réaliser ces dépistages. Pour rappel,

la commission ? L'amendement n° 100 rectifié renvoie au décret le soin de préciser les situations dans lesquelles l'orthoptiste pourrait intervenir en accès direct avec moins de précisions et de critères que ce qui est prévu par l'article 40. La marge de manoeuvre du pouvoir réglementaire

à conditionner l'accès direct aux orthoptistes à la réalisation d'un bilan préalable par un ophtalmologiste datant de moins de trois ans. Pour autant, cette condition pourrait pénaliser l'accès aux soins visuels de certains patients résidant dans des zones fortement sous-dotées en ophtalmologistes. En outre, la précision introduite par l'Assemblée nationale permet déjà de garantir la réalisation d'un bilan visuel par un ophtalmologiste à chaque renouvellement de prescription de corrections optiques, que la prescription initiale ait été faite par un orthoptiste ou par un ophtalmologiste. L'amendement n° 730, quant à lui, conditionne

mais il maintient dans le même temps les conditions de la prescription médicale préalable, ce qui est contradictoire avec l'idée d'un accès direct dans les zones caractérisées par un manque d'ophtalmologistes. Comme le disait la présidente Catherine Deroche précédemment, je ne suis pas sûre que les orthoptistes aillent s'installer là où il n'y a pas d'ophtalmologistes. Ensuite, il est incorrect de dire que les orthoptistes exercent une activité médicale : ce sont des auxiliaires médicaux. À défaut d'un retrait, l'avis sera défavorable. n° 101 rectifié est restrictif dans les compétences que les orthoptistes pourraient exercer sans prescription initiale. Il empêcherait les bilans visuels et les primo-prescriptions de corrections optiques. Il est donc peu probable qu'il permette de pallier les difficultés d'accès aux soins visuels, auxquelles l'article 40 entend répondre. Par ailleurs, la disposition introduite par l'Assemblée nationale visant à exiger qu'un bilan visuel préalable soit réalisé par un ophtalmologiste

n° 733 a pour objet la suppression de la possibilité pour les orthoptistes de prescrire des lentilles de contact à leurs patients. Les orthoptistes peuvent déjà adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. Il n'y a donc pas de raison de les en empêcher dans le cadre d'un accès direct. C'est une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable.

L'amendement n° 188 de la commission vise précisément à prévoir que les bilans visuels réalisés en accès direct par les orthoptistes seront soumis à des critères d'âge définis par décret, après avis du Conseil national professionnel d'ophtalmologie. La loi n'est pas la mieux placée pour définir ces critères d'âge. Par ailleurs, l'amendement ajoute beaucoup de complexité aux modalités de réalisation des bilans visuels par les orthoptistes en prévoyant des bilans préalables par un ophtalmologiste, avec des anciennetés variables en fonction de l'âge du patient. De telles rigidités me semblent incompatibles avec l'exigence de fluidité de l'accès aux soins visuels. À défaut d'un retrait, l'avis sera défavorable.

j'ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, de M. Gudni Johannesson, président de la République d'Islande. Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt et à la sympathie qu'il porte à notre institution. M. Johannesson est accompagné par Mme Françoise Gatel, présidente déléguée pour l'Islande du groupe d'amitié France-Europe du Nord. Après avoir participé à un séminaire sur l'hydrogène vert, organisé par le groupe d'amitié, présidé par notre collègue, M. André Gattolin, il s'est entretenu avec M. Roger Karoutchi, vice-président du Sénat. Au nom du Sénat de la République, je lui souhaite la bienvenue et je forme des voeux pour que son séjour en France contribue à renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays. Nous

Merci

le protocole de renouvellement optique, dit Rottier, qui permet la réalisation par l'orthoptiste d'un bilan visuel assez complet ; le protocole de rétinographie non mydriatique, dit Muraine ; ou encore le protocole de dépistage de la rétinopathie diabétique. La précision prévue dans cet amendement n'apporterait donc pas de valeur ajoutée. On peut considérer qu'il est presque satisfait, au regard de ce qui existe déjà et de ce qu'il est possible de faire en matière de coopération dans la filière visuelle. C'est une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable.

à Mme Florence Lassarade. L'article 41 du projet de loi revient sur une avancée introduite par le Sénat dans la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, qui rend effective la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes d'adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales datant de moins d'un an. Cet article restreindrait les conditions de renouvellement des prescriptions par par un kiné en renvoyant aux partenaires conventionnels le soin d'en définir les modalités de prise en charge financière. Il s'agit de limiter le champ d'application de l'alinéa 9 de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique en donnant la main aux seuls partenaires conventionnels pour en dessiner les contours.

La possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes d'adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales datant de moins d'un an est ainsi pleinement et directement applicable depuis le 28 avril 2021, contrairement à ce que suggère l'exposé des motifs du PLFSS. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer cet article.

aux masseurs-kinésithérapeutes d'adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. Toutefois, cinq ans après la loi, le décret d'application censé préciser les conditions de prise en charge des actes prescrits dans le cadre de ces renouvellements n'est toujours pas paru. C'est la raison pour laquelle le Sénat avait supprimé la nécessité de ce décret dans la loi Rist. Néanmoins, pour que ces renouvellements soient possibles, il faut que l'assurance maladie en détermine les conditions de prise en charge, dans un cadre conventionnel, avec les représentants des masseurs-kinésithérapeutes. C'est précisément l'objet de cet article 41. Pour être cohérente, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut,

qui s'ajoutent ainsi aux 9,3 millions de personnes vivant déjà en dessous du seuil de pauvreté monétaire, il semble plus que jamais nécessaire de faciliter l'accès à la santé de tous nos concitoyens. Alors que la protection de la santé est inscrite dans le préambule de la Constitution, que le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite quels que soient ses revenus, une médecine à deux vitesses continue à progresser, favorisant les favorisant les personnes qui peuvent assumer les dépassements d'honoraires aux dépens des autres. C'est ainsi que se crée une véritable fracture dans l'accès aux soins, au détriment des Français les plus modestes. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise donc à encadrer cette pratique des dépassements à 50 % du tarif opposable, tout en étudiant l'opportunité d'une revalorisation tarifaire des prestations techniques et cliniques pour une plus juste rémunération des actes des professionnels de santé. J'ajoute que, selon la Drees, en 2018, les 10 % des habitants les mieux lotis ont une accessibilité au système de soins six à huit fois supérieure à celle des 10 % des habitants

La loi prévoit aujourd'hui que les dépassements d'honoraires excédant « le tact et la mesure » sont sanctionnés. Cette disposition permet d'adapter le régime de sanctions selon les situations. Un décret prévoit ainsi que le tact et la mesure s'apprécient en fonction de la complexité de l'acte réalisé, du temps consacré, du service rendu au patient, de la notoriété du praticien, etc. Prévoir un pourcentage de dépassement d'honoraires serait, au contraire, une mesure peut-être trop rigide qui induirait une systématisation. Pour ces raisons, c'est une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Avis

entre les médecins et l'assurance maladie, sur la contribution des médecins à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins. Devant le défi que représente la désertification médicale de certains territoires, il apparaît cohérent que la convention médicale se saisisse de cette question dans son processus de négociation multipartite. Il s'agit non pas d'envisager le conventionnement sélectif ou tout dispositif coercitif, mais de faire en sorte que les médecins puissent, dans leur espace de discussion avec l'assurance maladie, se saisir de la question de l'offre de soins sur le territoire. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement l'avis de la commission ? L'amendement prévoit que la convention médicale détermine la participation des médecins à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins. Ces dispositions ont été adoptées en 2019 dans le cadre de la loi Santé. L'amendement est donc satisfait par le droit en vigueur. C'est donc une demande de retrait, ou, à défaut un avis défavorable.

ainsi que les étudiants achevant leurs études de médecine, à réaliser des remplacements ou à effectuer un exercice salarié en cabinet libéral dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. La majorité des nouveaux médecins commencent en effet leur carrière par des remplacements : la mesure envisagée dans cet amendement permettrait alors de les encourager à réaliser ces premiers remplacements dans les zones sous-dotées en médecins.

en 2018 avec, respectivement pour ces deux régions, environ 15 % et 12 % de personnes vivant en zone sous-dense. C'est le cas de 1,8 million de personnes en Île-de-France. Ainsi, près d'un Français de plus de 18 ans sur dix n'a pas de médecin traitant ; l'UFC-Que Choisir estimait en 2019 à 44 % la proportion de médecins qui ne peuvent plus accepter de nouveaux patients. Cela constitue une perte de chance et une inégalité grave dans l'accès aux soins.

de former de futurs médecins, ainsi que dans une politique de relance des services publics de proximité. Il est effectivement très difficile de demander à de jeunes médecins qui commencent leur carrière d'aller vivre dans des zones dépourvues de services publics et d'infrastructures attractives ; c'est vrai pour toutes et tous. L'installation est déjà régulée pour les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les kinés et les infirmières.

concomitante avec la cessation d'activité libérale d'un médecin exerçant dans la même zone. Nous avons conscience que cette mesure ne réglera pas tout, loin de là, mais elle s'inscrit dans une démarche de régulation des médecins d'exercice libéral,

où l'exercice salarié et l'absence de dépassement d'honoraires sont la norme. Ce mode de fonctionnement concilie parfaitement, à mes yeux, les aspirations des médecins et la préservation de l'accès aux soins de proximité. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est l'une des mesures importantes qu'il

ils doivent patienter pendant des mois avant de consulter un médecin spécialiste et parviennent de plus en plus difficilement à accéder à un médecin généraliste. Pour répondre à cette difficulté, le présent amendement vise à mettre en place

L'État et les collectivités locales financent depuis de nombreuses années des mesures incitatives à l'installation de médecins en zones sous-dotées, sans résultat probant. L'extension des déserts médicaux témoigne donc clairement de l'inefficacité des actions mises en oeuvre jusqu'à présent. Nous devons aujourd'hui instaurer des règles de régulation territoriale pour l'installation des médecins, comme il en existe déjà pour de nombreuses autres professions de santé.

Le principe de la liberté d'installation demeurera, mais le conventionnement ne sera possible que de manière sélective pour les nouvelles installations. Il nous faut désormais effectuer des choix clairs en matière de lutte contre la désertification médicale, afin de garantir l'équité d'accès aux soins pour l'ensemble de nos concitoyens, en tous points du territoire.

conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de l'exercice professionnel des médecins et à leur formation. La voie de la régulation

le présent amendement, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que dans des zones définies par les ARS, en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l'assurance maladie d'un médecin s'installant en zone surdense conclu que dans le cas où un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d'installation, mais instaurerait un conventionnement territorialisé. Nous prévoyons également une évaluation de ce dispositif,

En l'absence de telles clauses, le conventionnement des jeunes médecins serait conditionné à l'exercice de leur activité au moins un jour par semaine dans une zone sous-dotée en offre de soins.

sur ce sujet -, l'obligation pour la convention médicale de déterminer les modalités de participation des médecins à la réduction des inégalités dans l'offre de soins. En revanche, le Sénat avait rejeté un dispositif de conventionnement sélectif dans les zones surdotées.

un médecin s'étant vu refuser son conventionnement en zone surdense n'irait pas nécessairement s'installer là où sa présence est la plus nécessaire. En outre, l'obligation d'exercer un jour par semaine, pendant cinq ans, en zone sous-dotée, qui est proposée dans les amendements n 642

avec plus de 15 000 médecins maîtres de stage universitaire de deuxième et troisième cycles ; le développement de l'exercice coordonné ; le déploiement des assistants médicaux, avec plus de 1 500 contrats signés, dont 54 % en zones sous-denses ; et la signature des premiers contrats de début d'exercice, pour inciter les jeunes médecins et les remplaçants à exercer dans les zones sous-denses.

À chaque fois que j'ai abordé ce sujet avec vous, vous avez été à mon écoute, je tiens à le dire dans cet hémicycle. Merci donc pour cette bonne nouvelle ...